Si la problématique actuelle est plus à la gestion des retours de jeunes partis faire le djihad, il convient de modifier les conditions de l'autorisation de sortie du territoire des mineurs, que nous avons rétablie dans la loi de 2016. Ce rétablissement avait pour objet de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l'organisation dite de « l'État islamique ». En effet, selon le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces Français, essentiellement des jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350. Ce même rapport note d'ailleurs que « les départs de jeunes Français vers la Syrie n'ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s'est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d'opérations la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s'y opposer ». La volonté du législateur- c'est le fond du sujet

par « un contexte international marqué par le départ de Français- dont certains mineurs -sur des théâtres d'opérations de groupements terroristes ». Or l'application de ce nouveau dispositif prévoit que l'AST soit matérialisée par la présentation d'un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national, accompagné de la copie de la pièce d'identité du titulaire de l'autorité parentale. Autant dire Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n'aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d'identité de l'un de ses parents afin de remplir l'ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d'emprisonnement et des amendes pour fausse déclaration qui le dissuaderont. Il n'y a donc aucun contrôle dans les mairies, comme cela se faisait jusqu'en 2013. Dans cette affaire, il convient de protéger l'enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations. Aussi, afin de rendre réellement efficace l'AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence pour les sorties individuelles, selon des modalités à préciser par voie réglementaire. Je demande simplement au Gouvernement que l'on respecte la loi qui a été adoptée par le Parlement.

Ce serait une charge nouvelle forte pour les communes, qui vont devoir acheter des tampons, divers papiers,

Je constate que M. Grand a un certain nombre d'idées à soumettre, mais j'attendrai d'en avoir pris plus amplement connaissance,

la disposition législative ne soit privée de son effet utile par des dispositions réglementaires insuffisantes. Je remercie notre collègue Jean-Pierre Grand

cet amendement est essentiel. Je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. J'ai bien compris que M. le ministre d'État souhaitait attendre, mais, pour ma part, j'accorde vraiment beaucoup d'importance à la mise en oeuvre

Nous sommes dans un espace ouvert où, sans autorisation de sortie du territoire, un mineur peut sortir du territoire national et quitter l'espace Schengen sans autorisation. Responsabiliser les parents,

vaut pour les mairies correctement tenues, mais je suppose que la vôtre l'est également ... Concernant l'achat des tampons, monsieur le

Nathalie Goulet, pour explication de vote.

monsieur le ministre

M. David Rachline. Cet amendement vise à rendre automatique l'expulsion d'un étranger coupable d'actes de terrorisme tels que définis à l'article 421-1 du code pénal. Actuellement, l'expulsion est une peine complémentaire et facultative soumise à une durée maximale de dix ans d'interdiction du territoire. Lorsqu'un étranger trouble gravement l'ordre public par le vecteur le plus lâche qui soit, le terrorisme, il rompt à jamais le lien de confiance que la France lui avait donné. Il n'y a plus aucune raison qu'il bénéficie à nouveau de l'accueil

de la commission ? Cet amendement, qui vise à rendre obligatoire le prononcé d'une peine complémentaire, est inconstitutionnel. D'ailleurs, son auteur le sait parfaitement. Il faut toujours prévoir la possibilité pour le juge

l'avis de la commission. Comme vous le savez, le principe constitutionnel d'individualisation des peines, garanti par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,

Cet article vise à transposer dans notre droit commun le régime des perquisitions administratives de l'état d'urgence, à cela près qu'il s'agit non plus de « perquisitions » mais de « visites », qui pourront toujours se faire sur la base de simples suspicions et sur des critères extensifs et imprécis. La différence réside également pour le Gouvernement dans l'introduction d'une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de Paris, communiquée au parquet de Paris. cela ne constitue en rien une garantie. Soumis à la pression et contraints de travailler dans l'urgence et en petit nombre, ces magistrats se verront difficilement refuser ce genre d'intervention. En outre, comme le soulève le Syndicat de la magistrature, le texte ne prévoit pas quelles pièces seront versées au dossier qui lui sera soumis, et l'appréciation de l'autorité administrative résultera des éléments fournis par les services de renseignement. Encore une fois, si la commission des lois propose avec prudence de convoquer de nouveau le Parlement en 2021 pour s'assurer de l'efficacité de telles mesures, nous refusons, pour notre part, leur inscription dans notre droit commun, et ce pour quelque durée que ce soit. Mes chers collègues, ne déshonorons pas notre rôle de défenseurs des libertés individuelles en faisant montre de tolérance avec ce genre de mesures largement attentatoires à nos droits et libertés fondamentaux

de l'article 4. Nous considérons que nous sommes allés assez loin dans toutes les mesures possibles, notamment en matière judiciaire

équilibre. Vous avez été sensible au fait que, à Paris, où il y a le procureur chargé sur l'ensemble du territoire national de la lutte contre le terrorisme,

administratives contrôlées par le juge administratif à un système mi-judiciaire, mi-administratif. On ne comprend pas très bien dans quel sens tant la séparation des pouvoirs est nécessaire.

au sein duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne répondant aux mêmes critères- trop peu restrictifs -que ceux de l'article 3, toujours aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme. Nombreux sont, ici encore, les droits fondamentaux susceptibles d'être mis à mal par cette mesure par cette mesure : droit de propriété, inviolabilité du domicile, droit au respect de la vie privée et familiale ... Ici encore, les garanties apportées sont insuffisantes et le contrôle juridictionnel limité. Ce texte est vertigineux, mes chers collègues, et l'unanimisme qu'il recueille contre lui parmi les professionnels du droit et les institutions de défense des droits de l'homme semble impuissant à faire vaciller les certitudes qui animent le Gouvernement. de citer les mots très forts de Mireille Delmas-Marty, professeure émérite au Collège de France, dans sa lettre ouverte au Président de la République : « Il n'y a pas à choisir, monsieur le Président, la sécurité ou les libertés. Vous-même et votre gouvernement, sous le contrôle du nouveau Parlement, vous devez assurer l'une et l'autre, en acceptant qu'elles ne soient absolues ni l'une ni l'autre.

avoir lu l'oeuvre ! -rappelait la finitude humaine, il ne disait rien d'autre. Ce n'est pas en introduisant dans le droit de notre pays, après les réformes sécuritaires accumulées depuis la loi de novembre 2001, les principales dispositions qui accompagnent l'état d'urgence que vous vaincrez les fureurs sacrées du terrorisme radical. » Si ces mots ne peuvent vous convaincre, mes chers collègues, peut-être peuvent-ils vous faire réfléchir,

au risque de terrorisme, sans le droit d'assigner à résidence des personnes ou sans la possibilité de prendre une mesure administrative de perquisition sous le contrôle du juge ? Deux raisons

en dehors des grandes théories que l'on peut faire et que j'aime beaucoup- il n'y a pas de raison de s'en priver ! -, la lutte contre le terrorisme est aussi quelque chose de pratique et d'opérationnel. Il arrive que l'administration ait des renseignements qui proviennent soit d'une source étrangère soit d'une source nationale, mais qu'une seule personne ait à en connaître. Si on révèle l'information,

Il faut donc donner à l'administration le moyen de lever le doute : la perquisition peut être, dans ce cas, le moyen. Pour que cette perquisition puisse être admise, il faut qu'elle soit fortement

la plupart du temps, le procureur de Paris se saisira, il ouvrira une enquête préliminaire et on garantira l'efficacité de la procédure, parce qu'on sera dans le champ de l'investigation pénale. Cet article 4 encore que l'article 3, un leurre. Il s'agit de dire à nos concitoyens : nous nous libérons de l'état d'urgence, mais, soyez rassurés, nous inscrivons les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Eh bien moi, politiquement, cela me dérange

Parce qu'il faut, à un moment donné, sortir des mesures liées à l'état d'urgence et ne pas les verser dans le droit ordinaire, parce que, pour moi, les libertés fondamentales de notre République sont les valeurs essentielles nécessaires à l'exercice de la démocratie telle que nous la concevons,

Or si l'anonymat est garanti pour les agents effectuant la visite, dont seuls le service et la qualité figurent sur l'ordonnance, il ne l'est pas pour l'officier de police judiciaire présent sur les lieux. Ensuite, l'anonymat doit être garanti dans le procès-verbal de visite dressé immédiatement après les opérations, qui doit impérativement être signé par les agents y ayant procédé et par l'officier de police judiciaire présent.

pour certains actes de procédure pénale. En effet, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a instauré une procédure permettant à tout agent de police ou de gendarmerie nationale, dans certains cas et pour certains actes de procédure, d'être identifié

ne vise pas à faire application de l'ensemble de cette disposition, qui comporte de nombreuses conditions et garanties s'agissant de procédures pénales, mais à s'inspirer du dispositif d'identification qui y est mentionné, étant entendu que les procès-verbaux de visite, n'ayant pas le caractère d'actes de procédure pénale, n'ont pas à être entourés d'un formalisme identique.

L'article 4 du projet de loi permet de retenir la personne visée par la visite lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite. Cette retenue ne peut excéder quatre heures. Dans son texte initial, le Gouvernement avait prévu une simple information du juge des libertés et de la détention de Paris dans le cas où une personne ferait l'objet d'une telle retenue, à l'exception du cas des mineurs, devant donner lieu à un accord exprès de ce La commission des lois a étendu l'accord exprès du juge aux personnes majeures. Le Gouvernement estime qu'une telle procédure n'est pas nécessaire et souhaite en revenir au texte initial. En effet, la modification proposée par la commission serait lourde de contraintes, notamment lorsque les perquisitions se déroulent tôt le matin, ce qui est souvent le cas, et pourrait conduire, en cas de difficulté matérielle à obtenir l'accord du juge de manière immédiate, au départ de l'individu, qui serait particulièrement préjudiciable si la visite devait se révéler positive. Au surplus, le Conseil constitutionnel considère avec constance qu'une telle mesure n'a pas, compte tenu de sa brièveté, à être autorisée par l'autorité judiciaire, alors même qu'elle constitue une mesure privative de liberté. C'est d'ailleurs le cas des retenues administratives faisant suite à un contrôle d'identité, introduites par la loi du 3 juin 2016

introduit par la commission des lois : se rapportant aux règles relatives aux nullités en matière d'actes du juge d'instruction, il est sans aucun lien avec les visites ordonnées sur le fondement des dispositions de cet article, qui n'ont pas de caractère pénal.

Elle constitue la traduction de la règle :, en vertu de laquelle le plaideur ne peut pas agir selon plusieurs voies de droit pour porter un même litige devant des juridictions différentes. La Cour de cassation considère que cette limitation est applicable également pour les visites domiciliaires ordonnées par les juridictions judiciaires en matière non répressive, et pas seulement pour les actes pris en application du code de procédure pénale. pénale. Le nouvel article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, issu du présent projet de loi, prévoit que l'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris, d'appel de Paris, puis d'un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce dispositif assure un droit au recours effectif pour contester la décision de visite, ce qui rend inutile le renvoi à des règles de procédure pénale.

de la commission ? Le Gouvernement souhaite supprimer une précision ajoutée par la commission. Il considère que les visites ordonnées en application de l'article 4 n'ont pas de caractère pénal et n'appellent pas de mesures spécifiques.

C'est ce qui devrait se faire de manière générale pour être efficace, d'autant plus que si, à l'occasion d'une visite domiciliaire, c'est-à-dire d'une perquisition administrative, on découvre des infractions, il est indispensable de pouvoir tout de suite rentrer

le travail mené en commun par les services de police et de gendarmerie et les services de la justice, sous l'égide du procureur de la République, conduise à ne pas recourir à cet article, dont on vient, d'une certaine manière, de démontrer une nouvelle fois l'inutilité.

à instaurer des mesures de transparence, financières, mais aussi techniques, pour s'assurer que les associations qui prennent en main des jeunes pour les désembrigader, rétablir le lien citoyen et lutter contre la radicalisation ont un minimum de compétences et sont

Sont collectés au sein de ce fichier les coordonnées du voyageur, ses informations bancaires, ses itinéraires de voyage et son régime alimentaire. L'existence même de ce fichier pose plusieurs questions, notamment au sujet du respect de la vie privée de nos concitoyens.

À quand la mise en place d'une réflexion sur le contrôle des fichiers de renseignement ? La sécurité des données de nos concitoyens face aux pirates informatiques n'est pas toujours garantie, même dans nos administrations. Il y a deux semaines, des centrales nucléaires américaines ont vu leurs réseaux informatiques infiltrés. Les données des voyageurs conservées pendant cinq années, un laps de temps bien trop considérable, sont plus que vulnérables face à des toujours

éléments terroristes revient à retirer un peu de liberté à chacun de nos concitoyens pour des résultats qui n'en valent définitivement pas la peine.

sénatrice, nous avons besoin de cet article. Vous n'ignorez pas que nous sommes tenus à une obligation de transposer les directives de l'Union européenne

de nos services dans la lutte contre le terrorisme et contre les formes graves de criminalité. Je veux enfin rappeler que la directive PNR prévoit des conditions d'encadrement très strictes, visent à assurer un équilibre entre la recherche d'effectivité et la garantie des droits et libertés des citoyens. Parmi ces mesures figurent notamment la mise en place d'un délégué à la protection des données, l'interdiction de collecter des données dites « sensibles », l'anonymisation des données à caractère personnel collectées au bout de six mois, ainsi que la stricte limitation des personnes habilitées à en connaître.

Franchement, toutes les garanties ont été données. Le Parlement européen s'est véritablement fait violence pour finalement adopter

En ce sens, le PNR représente une avancée favorable, même si elle comprend aussi ses faiblesses. Notre collègue a rappelé les difficultés rencontrées avec la commission des libertés

de suivi des données des passagers aériens, le PNR, et adaptent le droit français au droit de l'Union européenne en la matière, permettant ainsi aux services de sécurité et de renseignement d'utiliser ces données pour diverses finalités, notamment la prévention et la détection des infractions terroristes. La transposition de la directive PNR dans le droit commun français, qui se substitue à l'actuel système API-PNR France », ne représente en aucun cas une solution efficace pour lutter contre les actes terroristes. Ces mesures sont largement contournables, dans la mesure où de potentiels terroristes seraient tout aussi bien capables d'entrer dans l'Union européenne et en France par d'autres moyens de transport que l'avion. Je tiens à rappeler que les mesures de collecte de données masquées ciblant l'ensemble des citoyens ne représentent jamais une réponse adéquate à la menace terroriste. Elles mobilisent des sommes non négligeables au détriment de moyens de lutte antiterroriste plus efficaces. Surtout, ces mesures sont en opposition avec le principe de l'État de droit. En 2014 déjà, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé dans la directive de 2006 sur la rétention des données, jugeant disproportionnées la collecte et la conservation massives de données de citoyens qui ne sont suspectés d'aucun délit.

complémentaires en matière de police et de justice, est de nature à régler les problèmes que cette nouvelle législation vise à résoudre. Tel n'est pas le cas du trafic passager au sein de l'Union européenne.

Il était évidemment fondamental d'inscrire le PNR dans la présente loi. En effet, le cadre législatif français était jusqu'ici défini par la loi de programmation militaire de 2013, qui avait autorisé la création d'un fichier de passagers du transport aérien à titre expérimental jusqu'à la fin de L'Union européenne a mis beaucoup trop de temps à légiférer en la matière, puisque ce n'est qu'en 2016 qu'une directive a, enfin, obligé l'ensemble des États membres à se doter d'un tel fichier et à partager leurs informations avec leurs partenaires européens. Je veux surtout souligner l'extrême importance de la coopération internationale en la matière. Rien ne sert de créer un fichier sur les informations des voyageurs s'il n'est pas partagé à l'international. La coopération européenne est fondamentale, comme je l'ai encore souligné tout récemment dans une communication devant la commission des affaires européennes au sujet de la coopération européenne en matière de renseignement. Néanmoins, cette coopération européenne est loin d'être suffisante. J'ai été rapporteur d'un texte organisant la coopération en matière de renseignement avec les États-Unis contre la criminalité grave et le terrorisme. Il nous faut absolument mettre en place des cadres d'échange hors de l'Union européenne et hors de l'OTAN, notamment avec les pays se situant de l'autre côté de la Méditerranée. Ces pays sont eux aussi très concernés par le terrorisme et n'ont pas toujours les moyens de mettre en place des dispositifs aussi performants que les nôtres. L'échange d'informations doit aller de pair avec la formation. Nous avons là une vraie responsabilité. Le projet de loi autorise également la création d'un PNR maritime, ce qui est pertinent, mais insuffisant. Il faut là encore encourager et organiser la coopération européenne et internationale Aujourd'hui, en Europe, seuls le Royaume-Uni, l'Espagne, la Finlande, le Danemark et la Belgique disposent de dispositifs minimums dans ce domaine. Il faut pousser les États à aller plus loin et surtout impliquer tous nos autres partenaires européens. Il faudra aussi travailler sur notre cadre légal interne,

En effet, la mise en oeuvre de ce PNR fait encore l'objet de réflexions de la part du Gouvernement, s'agissant notamment des modalités de consultation des données qui seront collectées à ce titre. Une réflexion est

propre service de sécurité. Actuellement, cela leur est interdit au motif qu'ils ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés. Heureusement ! Les établissements publics

peuvent créer un service interne de sécurité pour exercer des fonctions de surveillance et de gardiennage en régie sans recourir au service de sociétés de sécurité privée. L'amendement vise à élargir cette possibilité aux personnes morales de droit privé à but non lucratif gérant des établissements de santé sociaux et médico-sociaux.

le secteur de la culture, dont l'activité pourrait tout autant justifier l'existence de ce type de service interne de sécurité, en particulier s'agissant des musées. Avant d'être envisagée, une telle évolution doit donc faire l'objet d'une réflexion plus large, à laquelle le Gouvernement n'est pas opposé, qui serait menée en concertation à la fois avec les donneurs d'ordre potentiels non inscrits au registre du commerce et des sociétés et avec le secteur de la sécurité privée, dont les équilibres économiques s'en trouveraient modifiés. Il convient néanmoins de souligner que les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, qu'ils soient publics ou privés, à but lucratif ou non,

privés médico-sociaux de créer leurs propres services. C'est cela l'objectif. Cependant, si l'on ne traite que les établissements sociaux ou médico-sociaux, on va laisser de côté d'autres établissements à but non lucratif, culturels ou autres, où la même question se posera. Le Gouvernement, monsieur le ministre d'État, peut-il prendre des engagements de calendrier ?

On me dit que la réflexion est en cours. Nous aurons des éléments à la fin de l'année.

C'est une évolution ambivalente puisque, d'un côté, elle permet de faire entrer dans la légalité des pratiques de renseignement et, de l'autre, elle révèle l'ampleur des méthodes techniques à disposition de nos services, au point de se demander parfois ce qu'il reste de notre vie privée et du secret de nos correspondances. Dans le contexte sécuritaire actuel, dont on nous a répété la gravité à maintes reprises, il n'est pas question de s'opposer à ce que nos services disposent de tous les moyens existants pour déjouer des attaques terroristes. dès lors que la loi dispose pour l'avenir, un contrôle minimal de ces pratiques doit être assuré afin que ces moyens ne soient pas utilisés à mauvais escient, demain et après-demain, une fois que la menace terroriste aura peut-être disparu. L'ancienne commission de contrôle, créée en 1991, a été remplacée en 2015 par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui dispose de pouvoirs un peu plus importants. Compte tenu du nombre d'outils techniques de renseignement, il semblerait utile d'étendre encore les pouvoirs de cette commission en lui donnant la possibilité de suspendre certaines opérations de renseignement pratiquées par certains services après avoir constaté des enfreintes

autorité qu'elle n'a pas. Cette autorité administrative indépendante dispose d'un pouvoir d'avis et de recommandation. Elle peut recommander au Premier ministre de prendre telle ou telle mesure. Si sa demande n'est pas suivie d'effet, elle peut saisir le juge, mais elle ne peut elle-même ordonner la suspension d'une opération. Seule l'autorité administrative dont dépend ce service peut le faire ou le juge.

Comme vient de le dire Michel Mercier, la CNCTR constate que la loi n'est pas appliquée correctement. Elle peut ensuite adresser une recommandation tendant à ce que la mise en oeuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits. Si le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites données lui semblent insuffisantes, la CNCTR peut saisir le Conseil d'État.

instaurent un nouveau régime légal de surveillance des communications hertziennes afin de tirer les conséquences de la question prioritaire qui a censuré les dispositions de l'article L.811-5 du code de la sécurité intérieure introduisant des mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne. Nous sommes inquiets de voir que l'article 8 élargit le champ des techniques de renseignement prévues par la loi du 24 juillet 2015. En effet, le recours à des techniques intrusives ne se limite pas à la prévention des actes terroristes. En raison de sa définition vague des « intérêts nationaux et de « l'ingérence étrangère », cet article permet également de viser des personnes en raison de leur militantisme réel ou supposé. En outre, l'absence d'un véritable contrôle juridictionnel préalable par une autorité indépendante laisse à l'exécutif toute latitude d'opération. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement n'émettant qu'un simple avis, le contrôle par le Conseil d'État n'est pas suffisant au regard de la nature de la mesure. Ensuite, un nouveau chapitre relatif à la surveillance de certaines communications hertziennes paraît destiné à la direction du renseignement militaire, sans aucune autorisation du Premier ministre ni avis de la Commission, qui se voit simplement « présenter » le champ et la nature des mesures prises. S'inspirant de la loi sur la surveillance des communications internationales de 2015, avec des durées de conservation des données disproportionnées- six ans et jusqu'à huit ans pour les données chiffrées ce chapitre n'offre aucune garantie à nos concitoyens sur le respect de leurs libertés fondamentales, pas plus que cette captation massive de données une avancée dans dans la lutte contre le terrorisme. Demandons-nous, chers collègues, ce qu'il adviendrait si nous gravions ces articles dans la loi, ce qu'ils permettraient aux mains d'un exécutif moins soucieux

de la commission ? Dans une décision du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a censuré le principe de l'« exception hertzienne », en vertu duquel la surveillance des communications empruntant la voie hertzienne était exclue de tout encadrement juridique et de tout système d'autorisation préalable. La censure de cette mesure sera effective le 31 décembre 2017. Il est donc essentiel de prendre position pour éviter tout vide juridique. C'est l'objet de cet article 8, qui vise à créer un nouveau cadre législatif

Cet amendement vise à réduire le champ de la collecte de renseignements, en supprimant de la liste le définissant « la prévention de la délinquance organisée ». La version actuelle de l'article 8 offre la possibilité de recourir à des interceptions de correspondances échangées par voie hertzienne pour lutter contre l'ensemble des infractions mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. Cet article renvoie à toutes les infractions suivantes : l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ; les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; la prévention du terrorisme ; la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Les auteurs de cet amendement considèrent que l'autorisation d'interceptions de ce type recouvre un champ trop vaste et proposent de le réduire.

Je voudrais rappeler que le régime hertzien allégé résiduel résultant des articles 8 et 9 du projet de loi concerne les communications diffusées sur les ondes, comme le sont les émissions de radio ou de télévision, que n'importe qui peut capter

correspondrait à ce titre au cas où une personne communiquerait publiquement. Il est donc clair que le fait de l'écouter n'attente en rien à ses droits et libertés. Or l'amendement n° 61 rectifié porte sur le régime du hertzien ouvert. Il vise à limiter le champ des finalités pour lesquelles ce régime peut être utilisé par les services de renseignement, alors que cette restriction ne serait pas applicable au hertzien privatif, qui constitue, lui, un régime intrusif. Par ailleurs, les communications hertziennes ouvertes, du fait de leur facilité d'utilisation et de la préservation de l'anonymat qu'elles permettent, sont assez prisées dans des activités

dans certaines régions du monde, la criminalité organisée représente un risque pour notre sécurité nationale de même nature que les risques souverains. Ainsi, la piraterie et l'industrie de l'enlèvement

qui définissent les modalités du contrôle assuré par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur les mesures de surveillance des communications hertziennes ouvertes mises en oeuvre par les services de renseignement. services de renseignement. Pour tirer les conséquences de la censure, le 21 octobre 2016, par le Conseil constitutionnel des dispositions instituant une « exception hertzienne », le Gouvernement a conçu un dispositif à deux composantes un régime de surveillance des communications hertziennes « privatives », c'est-à-dire assimilables à des communications échangées à titre confidentiel ou privé, titre confidentiel ou privé, qui constituera une nouvelle technique de recueil de renseignements et qui sera assorti de toutes les garanties prévues par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement en termes d'encadrement légal, notamment de prérogatives de contrôle reconnues à la CNCTR ; d'autre part, un régime hertzien allégé, résiduel, pour la surveillance des communications hertziennes ouvertes, c'est-à-dire des communications échangées sur un espace public et pouvant être interceptées par toute antenne placée sur leur « chemin », la CB, ou, par exemple. Il est essentiel que la différence entre ces deux régimes hertziens soit bien marquée, y compris en termes de contrôle par la CNCTR, dès lors que seule la surveillance des communications hertziennes privatives est susceptible de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances. À ce titre, pour le hertzien privatif, la CNCTR doit disposer de toutes les prérogatives de droit commun applicables aux techniques de renseignement. En revanche, pour le hertzien ouvert accessible aux services de renseignement, il faut qu'elle puisse s'assurer que ce nouveau régime ne sert pas à empiéter sur le champ des techniques de renseignement. Pour l'exercice de cette mission, il lui suffit d'avoir accès aux capacités d'interception, car elles sont spécifiques aux communications hertziennes ouvertes et permettent donc de vérifier qu'elles ne peuvent servir à d'autres utilisations. Le Gouvernement a cependant admis que la commission puisse aussi ponctuellement demander au Premier ministre un accès aux renseignements collectés et aux transcriptions et extractions pour s'assurer de cette absence de dévoiement. Il est donc proposé sur ce point d'en revenir à la rédaction du Gouvernement.

d'un autre point de vue et a, la semaine dernière, simplifié la procédure permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de recueillir les informations nécessaires à la conduite de sa mission de contrôle en supprimant la sollicitation préalable du Premier ministre. Bien que les surveillances mises en place au titre de l'« exception hertzienne » échappent à ce contrôle préalable, il lui est en effet apparu souhaitable de conférer à la CNCTR des pouvoirs de contrôle de même nature que dans le droit commun. C'est la raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable.

à rétablir le texte initial du projet de loi font totalement abstraction de la formulation élaborée par la commission des lois.

nous sommes dans ce cas précis. Enfin, elle est également chargée du contentieux de la légalité des autorisations de recours aux techniques de renseignement. Qu'il s'agisse de la décision du Conseil constitutionnel

s'agit de l'outil principal du contre-espionnage français. Nous avons une longue expérience,

nos services ont une mission de défense de nos intérêts nationaux, de prévention des risques pour notre souveraineté nationale et que et que l'exécutif de ce pays, Matignon, avec une longue tradition de responsabilité d'État, est en mesure de s'assurer que les services agissent de façon respectable, honorable. Je Je constate que le Conseil constitutionnel n'a pas émis d'autre exigence que celle d'un cadre légal minimal de ces interceptions.

il s'agit de donner à la Commission de contrôle des techniques de renseignement la possibilité de suspendre les opérations de recueil de renseignements par voie hertzienne encadrées par l'article 8. Quel

À l'article 8 du projet de loi, il est prévu la transmission à la délégation parlementaire au renseignement des recommandations et observations que la CNCTR juge nécessaire au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du chapitre V du code de la Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes ». Par coordination, nous proposons de retranscrire cette disposition dans l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, qui regroupe l'ensemble des dispositions législatives concernant cet organe parlementaire. Quel est l'avis de la commission

en mesure d'exercer son contrôle. Cet amendement étend donc les moyens de contrôle de la CNCTR sur les unités militaires opérant la surveillance de cette catégorie de communications.

la capacité d'écouter les transmissions radio entre deux avions qui approcheraient de notre espace aérien ou encore de surveiller des communications émanant d'embarcations qui seraient voisines du point de sortie d'un de nos sous-marins.

Je pense qu'il serait audacieux de prétendre que ces organismes se livrent à une vérification ponctuelle sur les interventions des services.

protéger la démocratie et sécuriser la vie de nos concitoyens.

autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières », tant dans la durée que dans l'espace. Ainsi, les contrôles concernant les titres autorisant le séjour pourront s'étendre jusqu'à 12 heures contre 6 heures aujourd'hui. Cette mesure est

un outil efficace tant pour les forces de l'ordre que pour les renseignements. En effet, force est de constater que les réseaux terroristes n'empruntent pas les chemins balisés par l'État et sont en mesure de déjouer ces contrôles généralisés, soit

ces mesures sont-elles destinées à empêcher la commission d'attentats terroristes ou à servir des politiques d'immigration toujours plus guidées par des objectifs chiffrés ? Alors que des attentats endeuillent régulièrement l'Europe, il nous paraît nécessaire de rappeler que, dans leur majorité, les sont citoyens des pays mêmes qu'ils visent. Les réseaux terroristes étrangers s'organisent à l'étranger et peuvent téléguider à distance des terroristes bien ancrés sur le territoire national. Sous cet angle, la question des contrôles aux frontières apparaît presque comme désuète. Mes chers collègues, cette vérité douloureuse doit nous servir à repenser les problématiques de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme sous un autre prisme que celui du contrôle de nos frontières et du tout-sécuritaire. La parole est à Mme Esther Benbassa, présenter l'amendement n° 30. L'objet de cet amendement est, une fois encore, de supprimer une disposition qui nous semble pour le moins En effet, l'article 10 laisse craindre, comme le dit le Défenseur des droits dans son avis du 7 juillet 2017, que, « en l'absence d'encadrement strict des conditions de mise en oeuvre des contrôles d'identité et et de garanties, de tels contrôles soient effectués de manière discriminatoire et/ou en vue de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées Cela dit, permettez-moi, mes chers collègues, une considération plus générale. Il est assez cocasse de voir le Sénat, qui a voté les textes les plus sécuritaires ces dernières années, se placer tout d'un coup en défenseur des libertés fondamentales. La commission des lois, par la voix de son rapporteur dont je salue le travail malgré nos différences de vues, a rendu le texte plus acceptable, au point que le Gouvernement a déposé de nombreux amendements pour rétablir son texte initial contre les quelques garanties apportées et

politicienne pour envisager les mesures dont nous débattons ici dans ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire le droit de demain et des générations qui viennent De nombreux attentats sont déjoués grâce au travail des services de renseignement, aidés des forces de l'ordre et de l'appareil judiciaire, mais il n'existe aucune loi à même d'assurer un risque zéro. Ne vous en déplaise, monsieur le ministre d'État, ne pas voter cette loi n'est pas avoir une responsabilité, si un attentat survient.

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement

En effet, l'expérimentation du port d'une caméra individuelle par les policiers et les gendarmes a été concluante : l'utilisation de ces caméras permet d'apaiser les tensions, de sécuriser les missions en limitant les risques de comportement agressif et d'apporter la preuve du bien-fondé d'une intervention. Ce qui a été concluant sur le domaine public le sera nécessairement sur le domaine public ferroviaire. Rappelons également que l'expérimentation opérée par les gendarmes et les policiers a duré deux ans seulement. La première année qui a suivi le vote de la loi relative à la sécurité dans les transports a été mise à profit pour effectuer des tests techniques au sein de la SNCF et travailler avec la police nationale sur le choix des matériels. La CNIL

des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à transmettre, en temps réel, les images captées par leurs caméras individuelles lorsqu'ils sont confrontés à une situation nécessitant l'appui de leur poste de commandement. Aujourd'hui, le dispositif autorisé par l'article L. 2251-4-1 du code des transports permet seulement aux agents qui en sont porteurs d'enregistrer leurs interventions. En cas d'incident effectif, le dispositif sert ensuite à collecter des éléments de preuve pour permettre le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs. En revanche, lorsque l'effet dissuasif du dispositif échoue, ce dernier ne présente aucune utilité pour assurer la sécurité des agents. Si les images étaient transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné, ce dernier pourrait conseiller les

disait : « Le code pénal tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l'administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes sans aucune discrimination, n'a aucun sens, ni en termes de principes, ni en termes d'efficacité. » Ces mots se voulaient raisonnables et rassurants. Ceux qui ont lu le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui savent que son contenu n'est, en revanche, ni raisonnable ni rassurant. Il y a quelques jours, le Parlement a voté une sixième prorogation de l'état d'urgence sans sourciller, comme à l'accoutumée. Soyons rassurés, cette prorogation sera la dernière, le président l'a promis J'ai cru un moment que M. Macron était un libéral à l'américaine, libéral économiquement et en matière sociale et sociétale. Je me suis trompée M. Macron n'est pas Obama, il est seulement libéral économiquement. Ce projet de loi bafouant les libertés individuelles et les fragiles équilibres qui fondent l'État de droit en témoigne. Avec ce texte, la société qu'on nous propose de construire n'est même pas une start-up, mais une société du soupçon permanent, laissée entre les mains des pouvoirs administratifs, où le préfet et le ministre de l'intérieur peuvent désormais remplacer Nous avons assisté à la dernière prorogation de l'état d'urgence. Une fois cette loi promulguée, nul besoin en effet de recourir à ce régime d'exception : il sera devenu notre droit commun !

Nous avons suivi attentivement ce débat et y avons participé. Je suis très

Le scrutin est ouvert.